quelle société voulons-nous incarner ? C'est à cette question que nous répondons ici. Car la manière dont une société traite ses animaux est le reflet des valeurs qu'elle se donne. Et, heureusement, ces valeurs changent ; elles vivent, elles évoluent. Aujourd'hui, l'animal sauvage n'est plus seulement une menace ou une proie. C'est un être sensible, qu'il faut protéger et respecter dans son intégrité. Notre rapport aux animaux sauvages a changé, et c'est heureux ! J'en suis convaincue, cette évolution est loin d'être anecdotique. C'est le témoignage d'un profond changement dans les mentalités, qui engage notre humanité et, plus profondément encore, notre dignité. En résumé, c'est la marque d'une société qui progresse, qui refuse de vivre dans le passé au nom de traditions qu'on ne pourrait pas questionner, uniquement parce qu'elles existent. C'est pour moi une fierté que les moyens d'améliorer le bien-être animal soient discutés ici aujourd'hui. Car la protection des animaux est évidemment un enjeu pour la biodiversité, mais c'est aussi un impératif moral. C'est une priorité du Gouvernement, en particulier C'est aussi une demande forte de la part de nos concitoyens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, 90 % des Français soutiennent la proposition de loi telle qu'elle a été déposée sur le bureau du Sénat. Les bases d'un large consensus politique sont là. La chose est assez rare en politique pour être soulignée. Et c'est logique, car nous sommes aujourd'hui mieux informés sur la manière dont les animaux ressentent leur environnement et nos interactions avec eux. Nous ne pouvons plus ni fermer les yeux ni détourner le regard. Aujourd'hui, j'en suis convaincue, l'heure de la responsabilité a sonné. C'est maintenant qu'il faut agir, au sein de cet hémicycle ! Vous le savez, le Gouvernement a pris ses responsabilités, à l'issue d'un travail de longue haleine, en formulant au mois septembre 2020 des propositions fortes, essentielles et audacieuses. D'abord, nous avons annoncé la fin progressive de la présence des animaux sauvages dans les cirques itinérants lorsque cette itinérance est incompatible avec le bien-être des animaux. Bien entendu, il ne s'agit pas de mettre en question l'attention que les circassiens portent à leurs animaux. Il s'agit d'acter collectivement qu'il n'est plus raisonnable de continuer à transporter des éléphants, des otaries ou des fauves de ville en ville. Aujourd'hui, combien de maires, de toutes tendances politiques, adoptent des arrêtés ou des voeux contre l'installation de ces cirques ? Comprenez-moi bien : de tels arrêtés sont illégaux, et ils ne font que renforcer les difficultés que la crise sanitaire a causées au monde du cirque. Mais c'est le signe d'une demande d'évolution qui parcourt notre société. Nos décisions ne sonnent pas, tant s'en faut, la fin des cirques. J'ai la conviction profonde qu'en aidant les circassiens à répondre à cette demande de changement, nous leur permettrons de pérenniser leur activité. Demain, les arts du cirque continueront de nous émerveiller et d'attirer tous les publics. Ensuite, il nous semble essentiel de mettre fin à la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums. Les études le montrent : ces animaux ont conscience de leur captivité, et ils vivent le delphinarium comme une prison. Nous avons donc annoncé la fermeture des deux delphinariums que compte notre pays, ainsi que l'interdiction de tout nouvel établissement. Enfin, nous défendons la fin des élevages de visons d'Amérique pour leur fourrure en France. Et je suis heureuse de voir que la commission des affaires économiques a maintenu cette disposition, tout comme je suis heureuse de voir que la société dans son ensemble évolue sur le sujet. La décision d'un très grand groupe de luxe français de ne plus recourir du tout à la fourrure est une bonne nouvelle. Nous avions annoncé aux professionnels une fermeture sous cinq ans, mais le débat parlementaire s'oriente vers une fermeture sous deux ans. Nous appliquerons bien entendu la date inscrite dans la loi, et nous avons d'ailleurs déjà obtenu, par la négociation, et en mettant en oeuvre les mesures de soutien appropriées, la fermeture de trois élevages sur les quatre que comptait notre pays. C'est, je crois, la preuve que nous sommes au rendez-vous quand il s'agit d'appliquer des décisions fortes, en travaillant étroitement avec les professionnels. À ce stade, en tant que parlementaires, vous avez deux options. La commission des affaires économiques a choisi de renvoyer au pouvoir réglementaire les décisions d'interdiction, ce qui était déjà possible, tout en en complexifiant les conditions. Je respecte cette approche, mais ma conviction est que nous devons soit laisser au pouvoir réglementaire suffisamment de latitude pour agir, soit inscrire directement dans la loi ces interdictions, comme l'ont souhaité les auteurs de la proposition de loi. Pour que le texte fasse concrètement progresser la condition animale dans notre pays, il est nécessaire d'agir vite, et d'agir dès aujourd'hui. Ce n'est plus le temps des demi-mesures ou, pis, des faux-semblants. Nos décisions doivent être fortes, ambitieuses, visionnaires, pour notre bien-être à nous et pour celui des animaux. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la direction dans laquelle je suis convaincue qu'il faut aller. Au milieu de ce grand tournant que prend notre pays, mon rôle, et celui du Gouvernement, est d'abord d'accompagner les professionnels concernés, d'avancer avec eux, non pas contre eux, de répondre à leurs inquiétudes en prenant le temps de les écouter et de les accompagner. C'est là mon devoir. Nous avons rencontré cette année, à nouveau, les représentants des établissements concernés. Il s'agit de femmes et d'hommes qui aiment leurs animaux. Pour ces personnes, c'est souvent plus qu'un métier ; c'est un mode de vie. Et je me suis engagée à être à leurs côtés dans ce mouvement, qu'ils ressentent comme un bouleversement. Former les professionnels à un nouveau métier, aider les entreprises à évoluer vers d'autres activités, trouver un refuge pour les animaux : sachez que, sur tous ces sujets, l'État sera au rendez-vous. au rendez-vous. Il n'est jamais facile de prendre de telles décisions. Créer un cadre ambitieux pour le bien-être animal est une réforme qui fera date ; c'est le marqueur d'un changement de société profond. Cette évolution, nos concitoyens l'attendent dès aujourd'hui. Ils la réclament. Ne reculons pas face à cette demande et à ce large consensus populaire. Le temps que nous prenons, c'est celui de la concertation et de la réflexion. On peut affiner, et évidemment débattre des propositions. C'est le rôle de la représentation nationale, et il me tient à coeur. Mais prendre des demi-mesures là où précisément des décisions fortes sont nécessaires est le meilleur moyen de manquer l'occasion et d'échouer à convertir l'essai. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont les yeux rivés sur nous pour que nous soyons capables de traduire dans la loi cette prise de conscience collective, avec responsabilité et ambition.

Dans ces pays, les règles relatives au bien-être animal sont plus développées que chez nous. La France ne peut plus rester à la traîne. L'appel auquel vous avez aujourd'hui à répondre est chaque jour plus fort. C'est, je pense, l'appel de notre époque, un appel pour plus de respect et de considération pour la nature qui nous entoure.

Monsieur le président, madame la ministre- chère Barbara -, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que la réflexion éthique autour du bien-être animal se construit depuis de nombreuses années, voire des décennies, la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie n'était, quant à elle, pas ou peu abordée dans les débats parlementaires. En tout état de cause, elle ne l'était pas de manière aussi volontariste et pertinente qu'aujourd'hui. Nous sommes en effet face à un débat de société majeur. Si le bien-être des animaux s'accompagne, la maltraitance, elle, doit être condamnée. C'est bien cela dont nous allons parler aujourd'hui, avec une volonté forte de sensibiliser, d'accompagner et de sanctionner lorsque c'est nécessaire. nécessaire. La maltraitance des animaux de compagnie est devenue une préoccupation majeure de nos concitoyens et un véritable enjeu de politique publique. Nous sommes en effet très nombreux Plus d'un foyer français sur deux détient un animal de compagnie, et une écrasante majorité de nos concitoyens attendent que nous allions plus loin sur ces questions. Il faut traiter une telle question- c'est aujourd'hui très attendu -, et en dépassant un certain nombre de clivages. Je me réjouis donc de constater que tous les parlementaires ont su se saisir du sujet et dépasser le registre de l'émotion pour proposer des solutions opérationnelles. Rappelons-le sans fausse modestie : la présente proposition de loi a été, certes, portée par la majorité présidentielle, mais construite initialement avec tous les groupes politiques. Vous connaissez dans cet hémicycle notre manière de faire les lois, avec une volonté toujours affichée : celle de la raison et du pragmatisme. Et je sais que votre chambre partage cette ambition de construire des dispositifs utiles et efficaces pour l'avenir. Nous aurons des discussions pendant cette séance, et certainement quelques désaccords à surmonter. Mais nous souhaitons, j'en suis sûr, avancer ensemble sur le sujet. J'ai fait de la maltraitance des animaux de compagnie un véritable combat. La première des maltraitances, c'est d'abord l'abandon. Un animal de compagnie n'est ni un jouet ni un consommable. Face à ce constat, le Gouvernement a la volonté d'agir concrètement. C'est d'ailleurs l'objet du plan d'action contre l'abandon des animaux de compagnie que le Gouvernement a lancé au mois de décembre dernier et qui trouve une résonance forte dans cette proposition de loi. Il s'agit de sensibiliser le grand public, d'accompagner les structures qui recueillent des animaux et de mieux sanctionner lorsque cela est nécessaire. Cette proposition de loi illustre le triptyque qui doit nous animer, je le crois, toutes et tous, pour mener un tel combat, avec des valeurs partagées : sensibiliser, accompagner et sanctionner.

Ils sont abandonnés sur la route des vacances, lors d'un déménagement ou dans d'autres endroits. Je le disais : un animal de compagnie, c'est une responsabilité. C'est bien en faveur de cette prise de conscience individuelle que nous devons collectivement oeuvrer. Cette future loi nous y conduira, notamment avec la création d'un certificat d'engagement et de connaissance préalable à l'acquisition d'un animal de compagnie ou d'un équidé. Si la responsabilité est bien individuelle, la lutte contre la maltraitance animale, notamment l'abandon des animaux de compagnie, est évidemment l'affaire de tous. C'est également au travers de l'amélioration des contrôles que nous trouverons des solutions efficaces. Nous aurons l'occasion d'y revenir en séance, notamment lors de l'examen du chapitre I concernant les ventes sur internet, que nous souhaitons profondément encadrer. J'aurai l'honneur de vous présenter, au nom du Gouvernement, des amendements auxquels je tiens particulièrement. tiens particulièrement. Le deuxième objectif est l'accompagnement. Il faut en effet accompagner ceux qui agissent. L'animal abandonné est souvent recueilli par des refuges, des associations, des familles d'accueil, qui font tous un travail formidable. Je tiens à saluer leur engagement au quotidien, souvent assuré par souvent assuré par des bénévoles. Je salue également l'engagement de nos élus locaux sur les territoires ou encore les services de fourrière. Je tiens également à saluer devant vous, et cela a une résonance toute particulière dans cet hémicycle, les professionnels de la santé des animaux que sont les vétérinaires, tous essentiels pour la mise en oeuvre des politiques publiques de lutte contre la maltraitance animale. C'est avec eux que nous devons construire l'ensemble des réponses à ces enjeux. J'ai beaucoup échangé avec tous ces acteurs depuis plus d'un an pour définir des mesures concrètes. C'est dans cette logique opérationnelle que le Gouvernement a réservé une enveloppe de 20 millions d'euros pour l'accompagnement des refuges au soutien des campagnes de stérilisation ou encore au soutien

Lutter contre l'abandon des animaux de compagnie, c'est en effet lutter plus efficacement contre des actes parfois odieux, également contre des sévices infligés à ces animaux de compagnie qui nous choquent tous et qui doivent être combattus avec force. Quelles qu'en soient les raisons, ce n'est pas acceptable ! Ce n'est pas la conception que nous avons tous du progrès ! La maltraitance doit être donc plus systématiquement et plus fermement condamnée. Je sais que vos propositions vont nous permettre de poursuivre dans cette voie.

Au-delà du domaine législatif, c'est aussi dans cet esprit de construction et d'amélioration continue qu'au sein du Gouvernement, nous avons souhaité mettre en place un observatoire de la protection animale des carnivores domestiques. Je m'y étais engagé à l'Assemblée nationale. Cet organisme a été installé au mois de

mes chers collègues, dans, Rudyard Kipling raconte l'histoire du « chat qui s'en va tout seul ». Derrière les facéties du félin, rétif à la domestication, on voit progressivement se tisser un lien fait d'intérêts mutuels et, bientôt, d'affection désintéressée. En fait, à travers son histoire, c'est l'histoire du lien homme-animal que Kipling nous décrit. « Le chat qui s'en va tout seul » : j'aime cette expression. Car l'ambivalence de la condition animale est résumée dans cette formule. Même quand il a un maître, l'animal a toujours cette part de mystère, d'inexplicable, qui fait qu'il ne lui appartiendra jamais tout à fait. Tout au long de mes travaux préparatoires sur cette proposition de loi, que j'ai entrepris dès le mois de février, j'ai gardé cette expression en tête. Elle m'a rappelé combien il faut aborder la question avec nuance, car l'animal est irréductible à ce que l'on voudrait qu'il soit et à ce que l'on projette en lui. Et je veux dire à quel point, au cours de mes travaux, j'ai voulu prendre la cause animale au sérieux. On a pu m'objecter qu'il y avait d'autres priorités, que nombre de nos congénères ne vivaient pas eux-mêmes dans une situation très enviable. Ce à quoi je réponds : est-ce une raison valable pour ne pas agir ? Cela fait des années qu'une proposition de loi sur les animaux de compagnie et sauvages n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour. Il faut saisir l'occasion de ce texte, qui traduit un désir d'évolutions législatives, après que l'animal a enfin été reconnu comme être sensible voilà cinq ans. On m'a objecté encore que la proposition de loi touchait un seul élevage de visons en France, quatre orques, cinq montreurs d'ours, vingt et un dauphins, une vingtaine de manèges à poneys, et, au total, pas plus de huit cents animaux sauvages dans les cirques. Ce à quoi je rétorque : et alors ? mes yeux, comme le soulignait le vétérinaire centenaire Michel Klein, récemment reçu et honoré par le président du Sénat, c'est aussi notre lien aux animaux qui nous « fait hommes ». La relation entre homme et animal est si ancienne qu'elle fait partie intégrante de notre condition humaine et de nos sociétés.

Un Français sur deux détient un ou plusieurs animaux. Et la façon dont nous abordons ces dispositions, qui, pour certaines, relèvent presque du cas particulier, a des effets en cascade sur la relation homme-animal en général. Pour autant, il faut se garder de voir dans cette proposition de loi l'alpha et l'oméga de la condition animale. Son périmètre est volontairement assez réduit pour permettre un travail approfondi dans le temps imparti. Il ne traite- et nous avons respecté ce périmètre -ni de chasse ni d'élevage professionnel. Ce n'est pas une loi « générale » sur les animaux, et la Constitution empêche de sortir du cadre du texte déposé sur le bureau de la première assemblée. Il y aura des déçus, non pas sur les objectifs, mais sur la méthode. Car il y a ceux qui suivent une éthique de la conviction et qui défendent des valeurs indépendamment des conséquences concrètes que leurs décisions peuvent avoir. Et il y a ceux qui défendent une éthique de la responsabilité qui s'attachent à ce que les conséquences pratiques de leurs actes soient le plus conforme possible à leurs valeurs. Avec la commission des affaires économiques, mon approche sur ce texte s'est située résolument dans une éthique de la responsabilité. Autrement dit, la commission a estimé qu'il y avait des idées intéressantes dans la loi : faire signer un certificat d'engagement et de connaissance pour toute première acquisition d'un animal, y compris de particulier à particulier, c'est symbolique, mais cela participe d'une bonne information. Nous nous sommes appuyés sur cette avancée pour voter en commission l'obligation d'attendre sept jours à partir de la signature du certificat avant d'acheter un animal de compagnie. Quand on s'engage pour une vie, on peut bien attendre une semaine. On peut acheter des animaux, mais ce ne sont pas des marchandises comme les autres. Je vous mets au défi de trouver meilleure idée pour lutter contre les achats d'impulsion Renforcer les sanctions pénales contre les actes de cruauté commis sur les animaux et contre les 100 000 abandons qui ont lieu chaque année en France était une nécessité symbolique et pratique. La commission a renforcé les sanctions contre la zoophilie en créant un délit d'atteintes sexuelles sur animaux, car les animaux ne peuvent jamais exprimer leur consentement. La commission a jugé qu'il y avait aussi de l'affichage, aboutissant à des articles peu opérationnels. des animaux dans les cirques sans s'interroger sur leur devenir et à l'interdiction de la reproduction des cétacés ; pour les vétérinaires, c'est un non-sens qui met en péril leur santé. Sur ces questions, nous préférons le dialogue avec toutes les parties prenantes pour parvenir à une sortie progressive des situations problématiques. Des questions se posent quelle alternative ? Va-t-on améliorer le bien-être de ces animaux s'ils sont vendus à l'étranger sans aucune garantie de contrôle ? Nous devons y répondre. C'est le rôle des conseils spécialisés que nous instituons. l'interdiction de vente de tous les animaux en animalerie, et pas seulement des chiens et des chats, dans une logique de prohibition. Pourtant, c'est le circuit le plus tracé, le plus surveillé et encadré. Il représente une part archiminoritaire des ventes de chiens et de chats, 20 000 achats par an pour 100 000 abandons. La commission a réautorisé ces ventes à la condition que leur encadrement soit renforcé et que la présence d'animaux soit interdite en vitrine. Elle s'est attaquée aux vrais trafics en renforçant la régulation d'internet et la lutte contre l'introduction illégale sur le territoire de 100 000 chiens et chats par an en renforçant les sanctions contre les fraudeurs. Je vous proposerai tout à l'heure un amendement important interdire la vente en ligne d'animaux de compagnie ailleurs que sur des sites agréés et responsables. À mon sens, c'est une avancée majeure. Parfois, la proposition transmise par l'Assemblée nationale traduisait une méconnaissance du terrain. pense d'abord à l'obligation de stérilisation des 10 millions de chats errants par les maires sans aucune compensation par l'État de la somme colossale que cela représente. Vous le comprendrez bien, le Sénat, maison des territoires, ne pouvait pas accepter que l'État se défausse ainsi de ses responsabilités. évoquer l'interdiction maladroite de l'activité des associations sans refuge, alors qu'il y en a plus de 3 200 en France et qu'elles réalisent un travail formidable pour pallier le manque de places en refuges. Soucieux de valoriser les bonnes volontés des acteurs de terrain tout en leur donnant un cadre, le Sénat a réautorisé ces associations sans refuge à confier des animaux à des familles d'accueil. Elles pourront récupérer des animaux de fourrière et présenter des animaux en animalerie pour les faire adopter. Pour résumer, j'approuve un grand nombre des articles du texte, mais je considère que certains d'entre eux relèvent de l'affichage politique. Je préfère valoriser des solutions opérationnelles, pratiques, scientifiques, et élaborées en lien avec les professionnels, les associations et les vétérinaires pour améliorer les conditions de vie de nos animaux. Dans la préparation de l'examen de ce texte, j'ai conduit plus de 50 auditions et effectué de nombreux déplacements, qui m'ont amenée à rencontrer des élus locaux, des inspecteurs vétérinaires, des associations et des professionnels formidables et passionnés. Je tiens d'ailleurs à les remercier chaleureusement de leur disponibilité et de la richesse de leurs témoignages. Les professionnels ont bien compris que la bonne application des lois votées était la condition pour que leur activité prospère. Charge à l'État d'en renforcer les moyens. L'appel à davantage de sensibilisation, de formation, de recherche sur les animaux est unanime. Nous avons voulu nous en faire l'écho en commission en instaurant, par exemple, une sensibilisation à l'éthique animale pour tous les élèves de France, de l'école primaire au lycée. À l'avenir, il faudra encourager ces vocations et valoriser ces compétences, en développant, par exemple, des formations en faune sauvage captive, aujourd'hui quasi inexistantes, dans les cursus vétérinaires. Améliorons encore nos pratiques, renforçons la qualité du lien entre animaux et humains, au lieu d'ériger des barrières qui nourriront à terme l'indifférence. Les animaux sont un enrichissement considérable et un réconfort pour nos vies humaines. Ils permettent un éveil qui réconcilie l'homme et la vie sauvage. Il faut des espèces protégées. Mais on ne peut pas sanctuariser la vie de l'ensemble des animaux au risque, sinon, de les sortir de nos vies. Si nous n'y veillons pas, c'est le conte de Kipling qui deviendra réalité. Il en ira de tous les animaux comme de ce « chat qui va tout seul ». On pourra alors dire d'eux, à regret : Il est le chat qui s'en va tout seul et tous lieux se valent pour lui. Alors, il s'en va par les chemins mouillés du bois sauvage, sous les arbres ou sur les toits, et tout seul. » Je suis saisi, par M.

permettez-moi tout d'abord de m'étonner de l'énergie contemporaine à mettre en place une écologie animale tandis que nous galvaudons l'écologie humaine au fur et à mesure des textes de bioéthique ! Je rappellerai néanmoins l'impératif pour notre civilisation de lutter contre la maltraitance animale, et pas seulement envers les animaux de compagnie. Nous sommes très sollicités par nos compatriotes sur ce sujet. Nous sommes ici pour répondre à leurs légitimes interrogations, voire inquiétudes. En 2021, la loi doit malheureusement pallier les carences éducatives, la montée de l'individualisme, le tout-consumérisme, l'hyperviolence, y compris envers la vie animale, et au défaut d'assimilation de certaines cultures importées sur notre sol vis-à-vis du respect animal. La loi doit notamment empêcher l'application d'autres lois sur notre territoire. Avant d'en arriver à ce stade, il apparaît déjà une dérive déontologique grave et un déficit démocratique dans notre assemblée quand la commission sénatoriale saisie au fond refuse que nous débattions de certains amendements et, donc, de certains sujets en invoquant l'article 45 de la Constitution. Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » Les amendements concernés visaient à supprimer l'abattage rituel et à imposer l'étiquetage automatique pour la bonne information du consommateur, afin d'inciter par la sélection dans les commerces à la pratique de modes d'abattage vertueux. La commission des affaires économiques et sa présidente Les Républicains ont accepté des amendements sur la détention d'équidés, sur les animaux de compagnie, sur les fourrières, sur les chats errants, sur l'interdiction de diffusion d'images d'animaux sauvages, et c'est heureux ! Mais elles refusent que nous discutions et adoptions un dispositif législatif sur l'abattage rituel. Ces amendements cosignés avec mon collègue Jean Louis Masson sont les seuls à avoir été censurés en commission, puis en séance. Cette irrecevabilité est éminemment politique et arbitraire, au point de rendre inconstitutionnelle la proposition de loi pour atteinte au bon respect de la procédure législative. Ma question est claire avez-vous peur de ce débat ? Avez-vous peur que ces amendements soient adoptés pour ainsi censurer l'opposition ? Y aurait-il une maltraitance positive ? Pour lutter contre la maltraitance animale, nous devons aborder trois domaines : les animaux de compagnie, la chasse et des animaux sauvages et, enfin, l'élevage.

Les amendements sur l'abattage rituel sont une nécessité, car il s'agit d'une crainte constante pour nos compatriotes, d'autant qu'un tel procédé est devenu ultramajoritaire dans certains abattoirs. La présidente de l'Association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité (Afaad) affirmait déjà en 2018 : « Les animaux de boucherie ont été les grands oubliés de la protection animale.

D'après le magazine spécialisé, le marché du halal représente 329 millions d'euros annuels en grandes et moyennes surfaces. L'institut Nielsen, spécialiste des études de consommation, a établi que les chiffres de vente ont augmenté de 65 % en en seulement cinq ans. « Alors que la demande en viande halal devrait correspondre à environ 10 % des abattages totaux, on estime que le volume d'abattage rituel atteint 40 % des abattages totaux pour les bovins et près de 60 % pour les ovins », Selon la Direction générale de l'alimentation (DGAL), le nombre d'animaux abattus selon un rituel religieux dépasse très largement les besoins intérieurs des minorités religieuses concernées.

Cette réalité caractérise une infraction manifeste et une violation du principe constitutionnel de liberté de conscience des consommateurs. Auteur du livre, paru aux éditions Presses de la Cité, Anne de Loisy juge que les chiffres que je vous ai cités seraient même sous-estimés. Elle C'est même la conviction d'un grand nombre des professionnels de la filière qui, sous couvert d'anonymat, s'accordent à dire que l'abattage rituel concernerait en fait 8 à 9 ovins sur 10 et au moins 5 bovins sur 10. » Les abattoirs sont donc complices de l'augmentation constante de l'abattage rituel, pourtant si décrié. Les consommateurs achètent de la viande abattue selon des normes religieuses qui leur sont étrangères sans en être informés. Je pense notamment à des produits transformés qui utilisent du minerai de viande. Venons-en à la pratique elle-même. L'abattage rituel est un acte de cruauté, qui interdit l'étourdissement préalable avant l'égorgement. Ainsi, l'animal agonise conscient sur le sol ; en témoigne le mouvement de pédalage de ses membres pendant de longs instants. En fonction des couteaux plus ou moins aiguisés et des exécutants plus ou moins barbares, l'abattage peut entraîner d'affreuses douleurs. L'animal agonise en attendant de longues minutes que le sang remplisse ses poumons et l'étouffe. L'acte est indigne d'une société civilisée.

que les militants extrémistes végans ne s'aventurent jamais dans ces abattoirs, préférant toujours s'attaquer violemment aux boucheries traditionnelles. Au-delà de la situation scandaleuse et officielle des abattoirs, les filières d'abattage clandestines se développent, dans les caves, dans les rues, au moment de la fête de l'Aïd-el-Kébir, dans de plus en plus de territoires de non-France où s'applique un droit de substitution : la charia islamique. Ces méthodes barbares, répétées impunément chaque année, sont un corollaire du désastre causé sur notre civilisation par l'immigration et l'islamisation de notre pays.

De son côté, la Fédération vétérinaire européenne (FVE) demande « l'étourdissement de tous les animaux, sans exception ». En tout état de cause, dans un État laïque, il n'y a pas de raison que, sous prétexte de préceptes religieux, l'on autorise une maltraitance inadmissible à l'égard des animaux et que l'on installe un séparatisme alimentaire dans les rayons des supermarchés, dans les cantines scolaires et dans les établissements publics. J'ai du mal à comprendre comment on peut vouloir interdire à un éléphant de réaliser des figures dans quelques cirques, mais passer sous silence l'abattage massif d'animaux agonisant pendant près de dix minutes avant de mourir. C'est faire preuve au mieux d'une hypocrisie, au pire d'une grande lâcheté. Nous aurions eu tant à proposer à ce sujet dresser un bilan des abus liés à l'abattage rituel des animaux de boucherie ; exiger la suppression de toute dérogation à l'obligation d'étourdissement préalable ; prendre des mesures pour un étiquetage spécifique, automatique et clair de la viande provenant d'un abattage rituel, de sorte que les consommateurs ne soient pas pris en otage à leur insu rendre publics les rapports réalisés lors des contrôles par les services de l'État et les dérogations pour l'abattage rituel accordées par le préfet. Il est temps de lever le voile sur ce qui se joue en catimini sur notre sol ! Mais tout cela est tellement scandaleux que vous préférez refuser d'en parler. Je veux rappeler à ceux qui auraient encore des étriqués que la Finlande, la Grèce, la Suisse, le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas interdisent totalement ces pratiques. Depuis 2015, l'article 515-14 de notre code civil proclame que les animaux sont « des êtres vivants doués de sensibilité ». Or force est de constater que cette affirmation de droit n'est pas suivie d'effet. La lutte contre la maltraitance animale, si elle n'est pas globale, est une mascarade

cette motion, vous vous rendriez complices, une fois de plus, de ces agissements insupportables et du délitement de nos institutions.

Plusieurs propositions de loi émanant de diverses tendances politiques sont à l'origine du texte que nous examinons aujourd'hui. Je ne doute pas qu'un très large consensus existe bien évidemment à l'encontre de la maltraitance animale. j'admets avec plus de réserves l'existence d'un consensus sur la définition même de la maltraitance. À écouter certains mouvements, tout animal domestique serait un animal maltraité en puissance ... Si nous voulons être sérieux, devons éviter tout raccourci. En effet, la réalité est bien plus complexe. L'histoire de l'humanité est intimement liée à celle de l'animal, et ce depuis des millénaires. L'animal est partie intégrante de notre condition d'homme. Ces relations doivent néanmoins être empreintes de respect et de dignité. La cruauté envers les animaux n'a pas sa place dans notre société ; elle constitue d'ailleurs un indicateur de son niveau de développement. de développement. Je me félicite que la commission ait renforcé les sanctions de plusieurs actes de maltraitance. Les sévices et les atteintes sexuelles sont ainsi plus lourdement punis. De nouvelles circonstances aggravantes ont été créées, afin de mieux protéger les animaux, ainsi que les enfants, lorsque ces actes sont malheureusement perpétrés sous leurs yeux. De même, la commission a intégré de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les trafics d'animaux. L'amende encourue est ainsi portée de 7 500 euros à 30 000 euros. Il était temps de rendre la sanction enfin dissuasive ! En dehors des actes de cruauté, la commission a sauvegardé le plus possible le principe de liberté ; nous le saluons. Ce texte Ce texte comportait initialement nombre d'interdictions qui satisfaisaient probablement certaines orthodoxies, mais qui demeuraient très éloignées de la réalité de terrain. Deux sujets me semblent bien illustrer ce point. L'interdiction générale de la détention d'animaux non domestiques dans les cirques et les delphinariums aurait eu un effet négatif sur la conservation des espèces et sur l'information du public. La solution retenue par la commission permet d'assurer la surveillance des cas de maltraitance, ainsi que leur sanction, y compris, le cas échéant, par la fermeture de l'établissement concerné. Dans la même logique, l'interdiction générale de la vente d'animaux par les animaleries ne résolvait pas les problèmes soulevés. Les animaleries dans notre pays sont professionnelles. Elles jouent un rôle important de responsabilisation, de sensibilisation et d'information du public. Plutôt que d'interdire purement et simplement une activité, nous préférons qu'elle soit encadrée et contrôlée, de sorte qu'elle puisse se dérouler dans des conditions satisfaisantes. C'est en renforçant la relation entre l'humain et l'animal que nous ferons reculer la maltraitance. La France détient aujourd'hui le triste record européen de l'abandon Ce fléau touche chaque année plus de 100 000 d'entre eux. Les animaux ne sont pas les égaux des humains, mais ils sont des êtres vivants, et non des jouets. Adopter un animal de compagnie n'est pas un acte anodin ; c'est un engagement dans la durée. Le certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce est une mesure essentielle

En renforçant la protection des animaux contre les actes de maltraitance et en améliorant l'information de nos concitoyens, la commission a su trouver les points d'équilibre dont le texte avait besoin. Notre groupe soutiendra l'adoption de la présente

alors que l'humanité est responsable de la sixième extinction de masse du vivant, il nous faut rompre avec cette conception dépassée selon laquelle la nature et les animaux seraient des objets et avec le mythe d'une humanité triomphante au-dessus de la nature. l'homme et l'animal sur un pied d'égalité, la frontière construite entre eux est artificielle et conceptuelle. Les études en éthologie le démontrent chaque jour. Oui, il est grand temps d'admettre que, dans notre société, la souffrance infligée aux animaux doit être pleinement prise en considération.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'est globalement satisfait du texte issu de l'Assemblée nationale, qui constituait une étape bienvenue dans la lutte contre la maltraitance et apportait une première série de mesures attendues par nos concitoyens, notamment sur l'amélioration des conditions de cession et de détention des animaux de compagnie, sur le renforcement des sanctions contre la maltraitance. Mais ce texte ayant un périmètre volontairement restreint, il est loin de s'attaquer à tous les aspects de la souffrance animale.

En revanche, il est tout à fait regrettable que, une fois de plus, le débat sur les pratiques cruelles de chasse nous soit refusé et soit absent d'un texte traitant notamment de tous les sévices que les humains font subir aux animaux dans le cadre de leurs divertissements. Mettre fin à la corrida, aux combats de coqs, à la chasse à courre ou encore au déterrage des blaireaux et des renards sont autant de combats qui demeurent d'actualité. Laissez-nous vivre ! Ce sont des pratiques d'un autre âge, que les Françaises et les Français rejettent dans leur écrasante majorité. J'en viens à l'examen du texte par la commission. Sous couvert d'une potentielle perte de lien entre les animaux et les humains, la commission a opéré d'importants reculs. Nous regrettons notamment qu'elle ait largement amoindri la portée de l'article 12, lequel ne prévoit plus l'interdiction progressive de l'acquisition, de la détention et de la reproduction d'animaux sauvages dans les delphinariums et les cirques itinérants. C'était pourtant l'une des mesures phares du texte. Il ne s'agit pas là de convictions personnelles. Les scientifiques sont unanimes. Comme le rappelle notre collègue Arnaud Bazin, il n'existe pas de mammifères non domestiques dont la physiologie et le comportement soient compatibles avec la vie dans un cirque itinérant ou un delphinarium. Nous regrettons également la marche arrière sur l'interdiction de la vente de chats et chiens en animalerie, qui était une demande forte des associations de protection animale et de nos concitoyens. revanche, nous nous sommes retrouvés sur plusieurs sujets, en particulier celui de la reconnaissance juridique des familles d'accueil d'animaux abandonnés. Ces dernières sont l'un des maillons essentiels qui, sur le terrain, permettent aux animaux de retrouver un foyer. Il est légitime de doter les associations sans refuge d'un véritable statut législatif. Nous saluons d'autres apports adoptés en commission, comme la création d'une circonstance aggravante pour les actes de cruauté sur un animal lorsqu'ils sont commis devant un mineur ou encore le renforcement des sanctions pour pénaliser drastiquement la zoophilie en France. France. L'obligation pour les maires de stériliser les chats errants a été abordée. L'État doit clairement engager des moyens supplémentaires pour soutenir les collectivités dans cet objectif de politique publique. Nous pourrons en débattre lors de l'examen du projet de loi de finances.

en faveur de la cause animale et d'une meilleure prise en compte des enjeux éthiques, écologiques et sanitaires. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires continuera à lutter contre la maltraitance animale, toute la maltraitance. La parole

les Français aiment les animaux. Ils les aiment tellement qu'ils en possèdent beaucoup : 15 millions de chats, 8 millions de chiens. Voilà des chiffres qui placent la France dans le peloton de tête européen aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie. Pourquoi un tel engouement ? Montée de l'individualisme ? Explosion des banlieues pavillonnaires ? Nouvelles formes de solitude ? Repli familial au détriment d'autres formes de sociabilité ? Quoi qu'il en soit, on observe une réciprocité accrue entre l'homme et l'animal. Nous ne pouvons que nous en réjouir, d'autant que cette évolution est récente. Il a fallu attendre 2015 pour que le Parlement reconnaisse aux animaux la qualité symbolique d'« êtres vivants doués de sensibilité Le texte qui nous est soumis aujourd'hui s'inscrit dans cette logique, au titre de laquelle le respect et la dignité de l'animal ne doivent pas se cantonner à de vaines paroles. Car beaucoup reste à faire. Nous aimons les animaux, mais nous les abandonnons aussi beaucoup. La France reste le pays d'Europe où l'on abandonne le plus d'animaux domestiques. Ils sont ainsi environ 200 000 par an à connaître ce sort. Et l'été 2021 ne les a pas épargnés, loin de là

Le texte proposé par les députés Loïc Dombreval, Laetitia Romeiro Dias et Dimitri Houbron entend remédier à cette crise de l'abandon, notamment par le biais du certificat de sensibilisation pour les futurs détenteurs d'animaux de compagnie.

commençant par l'épineux problème de la stérilisation des chats. Les associations de protection animale sont débordées par les abandons de chats. Or le contrôle des populations de chats errants sans propriétaire recouvre des enjeux de santé publique et de protection animale.

de « voeu pieux, mesure d'affichage au détriment des élus locaux [ ...] en l'état inacceptable ». Ces mots me paraissent quelque peu excessifs. Je partage pleinement les objectifs du rapporteur de l'Assemblée nationale. Il y a 10 millions de chats errants sur notre territoire. C'est surtout cela qui est inacceptable. Faute de moyens suffisants, l'obligation imposée ne pourra être pleinement assumée par tous les maires. Je rappelle que la stérilisation d'un seul chat coûte 120 euros. Dans mon département, la Drôme, certaines petites communes ne pourront pas assumer seules une telle charge. Enfin, il conviendrait d'opérer de manière simultanée sur les communes d'un même territoire pour que la stérilisation soit efficace. Je le sais, c'est un sujet prioritaire qu'il nous faudra résoudre rapidement. Mettons-nous autour d'une table- associations, parlementaires, maires, Gouvernement -, afin de réfléchir collectivement à une issue pérenne.

rapporteure a réécrit la disposition concernée en réintroduisant la vente d'animaux de compagnie, tout en incitant à la mise en place de partenariats entre refuges et animaleries. Cette réécriture va dans le bon sens, mais nous souhaitons aller plus loin. Nous proposerons que seuls les chiens et chats issus d'une association de protection des animaux ou d'un élevage puissent être autorisés à la vente. Enfin, je souhaite revenir sur l'article 12. Comme je l'ai indiqué, tout animal est un être sensible : le proclamer, c'est bien ; en tirer toutes les conséquences, c'est encore mieux. À ce titre, les animaux exhibés dans les cirques itinérants n'ont pas leur place dans des cages exiguës. Nous pouvons tous convenir que de telles conditions d'existence sont d'un autre âge. L'opinion publique en est consciente. Ainsi, il nous paraît cohérent d'en rester à la version de l'Assemblée nationale : interdire à terme la détention de la faune sauvage dans les cirques et les delphinariums. Sur ce sujet, nous ne partageons pas une vision trop timide et source de complexité. C'est pour notre groupe un vrai point de divergence.

À l'aube de la présidence française de l'Union européenne, notre main ne doit pas trembler. Il est nécessaire d'aller aussi loin que possible, mais avec méthode et concertation.

Certaines pratiques qui avaient cours jusqu'alors semblent aujourd'hui recueillir la désapprobation d'une majeure partie de la population. Je pense notamment à la fin des animaux non domestiques dans les cirques itinérants et les delphinariums ou à l'exploitation des animaux pour leur fourrure. est devenu un objet de consommation courante, abandonné à la moindre difficulté. Dès lors, c'est toute sa place dans notre société qu'il faut revoir. Les expositions au public pour inciter à l'achat sous le coup de l'émotion, l'élevage par des particuliers à des fins purement lucratives, la multiplication des annonces en ligne qui ne sont pas conformes à la loi, les interventions chirurgicales et esthétiques ... toutes ces pratiques persistent et nous poussent à faire évoluer le droit pour assurer, dans les textes et dans les faits, une meilleure protection des animaux. Le rapport remis au Gouvernement en 2020 par le député Loïc Dombreval était plus ambitieux que cette proposition de loi. Pour mieux protéger les 63 millions d'animaux de compagnie que compte notre pays, et pour mieux lutter contre l'abandon de 100 000 d'entre eux chaque année, notre collègue député a formulé 121 propositions. notamment la mise en place d'une attestation de connaissance obligatoire pour tout nouvel acquéreur, avec la création d'une formation en ligne, l'évaluation comportementale systématique des chiens à l'âge d'un an, l'interdiction des cessions de chiens et chats en dehors des refuges et des élevages avant l'âge de dix semaines, la limitation de la taille des élevages ou encore la mise en place d'un certificat de capacité pour tous les éleveurs. Les amendements que je défendrai au nom de mon groupe s'inspirent en partie de ce rapport et visent essentiellement à s'attaquer aux causes de l'abandon, en limitant les achats compulsifs. La réglementation et l'accroissement éventuel des contrôles sur les animaleries, ainsi que l'interdiction de placer les animaux en vitrine ne suffisent pas à répondre aux besoins des chiots et des chatons, qui doivent rester auprès de leur mère jusqu'à dix semaines au moins. Or les causes de l'abandon sont également liées aux problèmes comportementaux de certains animaux, parfois causés par une séparation précoce avec la mère. Je défendrai également des amendements concernant l'interdiction de la vente dans les animaleries. S'il est acceptable d'y trouver des poissons, les chiens et les chats n'y ont plus leur place. La loi doit l'indiquer clairement. Les conditions d'élevage des animaux de compagnie ont des conséquences non négligeables sur leur socialisation et donc sur leur futur comportement. Il convient de sensibiliser et de responsabiliser les particuliers en les incitant à recourir à l'adoption d'animaux abandonnés ou à se tourner vers des élevages respectueux du bien-être animal. nous nous réjouissons que la commission ait adopté notre amendement visant à mentionner, sur les offres de cessions d'animaux de compagnie, le nombre de portées de la femelle reproductrice au cours de l'année écoulée. Enfin, le coût que représente la détention d'un animal est loin d'être négligeable : frais vétérinaires, alimentation, maladies ... Il nous semble donc essentiel de mieux informer l'acquéreur au préalable.

Malheureusement, s'il va dans le bon sens, le renforcement des dispositions pénales ne changera pas la donne dans de nombreux cas. En effet, il n'est pas aisé de prouver l'élément intentionnel, par exemple dans le cas d'un abandon. De manière générale, nous aurions souhaité que la commission des affaires économiques aille plus loin sur un certain nombre de sujets. Les associations avaient déjà déploré le manque d'ambition du texte initial, et elles ont massivement exprimé, si l'on en juge par le nombre de messages reçus, leur désaccord vis-à-vis de certaines positions de la majorité sénatoriale.

Mieux informés sur les conditions de vie des animaux et les traitements qui leur sont infligés, les Françaises et les Français s'indignent, car ils aiment les animaux, et ils ont raison « l'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà ». En réalité, nous ne sommes pas encore parvenus à la question du bien-être animal. Nous n'en sommes qu'aux problématiques que pose la souffrance que nous infligeons aux animaux. Or, entre l'absence de souffrance et le bien-être, il y a tout un espace à conquérir. La majorité gouvernementale, qui a bien compris que le sujet avait pris une certaine importance dans notre société, nous soumet donc ce texte, une proposition de loi présentée par son groupe parlementaire et votée en janvier dernier à l'Assemblée nationale, après avoir esquissé quelques pistes dans la loi Égalim 1. initiale apportait des améliorations concernant le traitement des animaux domestiques. Ainsi, il interdisait les delphinariums et les spectacles d'animaux sauvages, ainsi que les élevages de visons.

de loi s'approche du seuil, mais ne le franchit pas. Ainsi, ses promoteurs ne se préoccupent que des animaux domestiques et de certains animaux sauvages. C'est déjà quelque chose, me répondra-t-on, mais, alors même que l'intitulé original, là aussi modifié par la commission- j'y reviendrai au cours des débats -, évoquait la lutte contre « la maltraitance animale », avec cet emploi du singulier qui suppose le général, toute une catégorie d'animaux en est absente, rayée du champ de vision.

mais, en divisant, on hiérarchise, et certaines catégories deviennent plus importantes que d'autres. Pourtant, les animaux victimes de l'élevage intensif, au-delà de leur situation, subissent aussi des actes de cruauté. Certains animaux mériteraient donc qu'on les protège de la maltraitance, et d'autres non En réalité, c'est la question du modèle de l'élevage intensif, soigneusement dissimulée pour que nous ne nous offusquions pas de ce système inhumain, qui se pose. Comment en sommes-nous arrivés à considérer que des êtres vivants et sensibles, capables de ressentir la douleur physique comme la souffrance psychique, ne méritaient pas un traitement digne ? Comment avons-nous pu organiser et systématiser de tels traitements, au nom du marché et du profit, en oubliant la nécessité de garantir une alimentation saine et durable à nos concitoyens, le bien-être à nos animaux, ainsi qu'aux personnes qui travaillent auprès d'eux, notamment les salariés des abattoirs, qui subissent la violence des cadences infernales et la déshumanisation de leur travail ? Au fond, le débat éthique sur la maltraitance animale devrait nous faire réfléchir à notre définition de l'espèce humaine,

et aux autres. Au V siècle avant notre ère, Pythagore affirmait déjà : « Aussi longtemps que les hommes massacreront des animaux, ils s'entretueront. En effet, celui qui sème les graines du meurtre et de la souffrance ne peut pas récolter la joie et l'amour ».

le développement de nombreuses associations de défense des animaux est une manifestation concrète de l'importance de la question du bien-être animal dans l'opinion publique. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous attendu par nos concitoyens pour arrêter la maltraitance faite aux animaux. En effet, un équilibre est ce titre, de saluer le travail de fond réalisé par notre collègue Anne Chain-Larché, d'une part, et par la présidente Sophie Primas, d'autre part, sur ce sujet très sensible, très humaniste, mais dont la dimension économique n'est pas négligeable. Aux côtés des animaux de compagnie, je veux évoquer les animaux de la ferme, dont nous ne parlons pas ce matin ; c'est d'ailleurs tout à fait légitime, car les éleveurs traitent correctement leurs bêtes et apportent un soin particulier et adapté aux différentes espèces. Les conditions de vie des animaux constituent désormais un sujet d'intérêt majeur et durable pour les citoyens-consommateurs, soucieux non seulement de la qualité des produits qu'ils consomment, mais également de leur mode de production.

C'est par cette approche globale et pluridisciplinaire que les éleveurs réussiront la transition vers un élevage plus durable. Il me semblait essentiel de le rappeler ici.

afin d'aider à la prise de conscience de ce qu'elle entraîne pour l'acheteur. Prendre le temps d'apprécier les contraintes que suscite l'adoption d'un chiot, d'un chaton ou d'un lapin est primordial avant toute transaction commerciale. Aussi, nous interdisons les pratiques inacceptables, comme le « satisfait ou remboursé » ou encore l'expédition postale. Les animaleries sont finalement au coeur de ce que nous voulons pour nos animaux de compagnie. Interdire les ventes dans les animaleries aurait conduit à un résultat très certainement inverse de celui qui est visé.

Les associations, aux côtés des élus locaux, accomplissent une formidable action quotidienne en faveur des animaux abandonnés. Reconnaissant leur travail immense, la commission a facilité et encadré le recours aux familles d'accueil, qui sont l'un des maillons de la chaîne permettant à ces animaux de retrouver un foyer.

mesure ayant évidemment un effet direct sur le bien-être animal. Autre avancée, nous avons alourdi les sanctions en cas de trafic et de vol d'animaux.

Une campagne nationale, dont les maires et les vétérinaires seraient les relais actifs, sera lancée pour rappeler l'intérêt de l'identification et de la stérilisation.

De plus, à l'heure du numérique, nous interdisons la détention et la diffusion de tout contenu zoopornographique et responsabilisons les moteurs de recherche. Une dimension préventive a été ajoutée à ce volet pénal les actions de sensibilisation à l'éthique animale et prévoyons la prise en charge précoce des enfants lorsque leur foyer a fait l'objet de signalements pour maltraitance animale. Enfin, s'agissant des animaux sauvages, il est permis aux delphinariums de poursuivre leur activité, moyennant la création d'un conseil spécialisé offrant une véritable expertise scientifique pour éclairer les décisions des pouvoirs publics dans le cadre de la recherche de solutions pour les cétacés. En cas de manquement constaté, des interdictions ciblées pourront être prononcées. Face aux critiques sur la santé des cétacés dans les parcs d'attractions- je pense aux lésions cutanées dues au chlore, au sonar des dauphins qui se réverbère sur les parois, aux bassins trop petits, etc. -, les pratiques évoluent. Le parc Astérix a annoncé, avant le dépôt de ce texte, la fin définitive de ses spectacles avec dauphins et otaries. Aujourd'hui, quelque 66 % des Français s'opposent à ces spectacles. Les exigences posées par le Sénat devraient permettre de contrôler le bien-être Dernier point important, la commission a voulu donner aux cirques les moyens d'évoluer en fixant une liste d'animaux autorisés. Les animaux sont véritablement doués de sensibilité- nous en sommes tous d'accord. Ce texte d'aboutir à une législation assurant leur protection et de faire de la lutte contre leur maltraitance une réalité. Les sénateurs s'apprêtent à durcir les sanctions, à responsabiliser les actes de vente et d'achat d'animaux, enfin, à mieux contrôler les liens entre animaux et humains.

En traduisant une partie des recommandations du rapport du député Loïc Dombreval sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés, cette proposition de loi a pour objet de répondre à une forte demande sociétale en ce qui concerne l'amélioration de la condition animale.

Comme sur la majorité des sujets sociétaux, les oppositions ont été fortes et les débats animés. La vitalité de notre démocratie passe aussi par ces échanges et ces réflexions sur la place et les droits des animaux. Toutefois, ne soyons pas dupes le dépôt de cette proposition de loi par la majorité présidentielle s'inscrit dans un calendrier électoral bien particulier, où la communication auprès des Français redevient importante. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des sujets sensibles, comme les conditions d'élevage ou certaines pratiques de chasse, a été volontairement mis de côté par l'exécutif et les parlementaires concernés. Dans ce contexte, et face à des questions sociétales qui intéressent les 50 % de Français disposant d'un animal de compagnie, et sûrement bien d'autres, nous ne devons pas tomber dans le dogmatisme et agir sans le concours du bon sens. Nous pouvons tous nous exprimer sur nos représentations du bien-être animal et débattre de nos solutions pour lutter contre la maltraitance animale. Notre expérience de parlementaires et nos différents vécus professionnels doivent nous servir à trouver des réponses à une problématique qui affecte et concerne bien des secteurs et des domaines d'activité. C'est la position que nous avons retenue au sein du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, position que nous défendrons lors de la présentation de nos différents amendements : pas de dogmatisme sectoriel, corporatiste ou même animaliste, mais simplement des solutions concrètes pour réellement lutter contre la maltraitance animale. Ce texte présente de texte présente de réelles avancées, qui feront sûrement consensus au sein de notre hémicycle. Je pense notamment à la création d'un certificat de connaissance pour les animaux de compagnie et les équidés, l'interdiction de la vente d'un animal de compagnie à un mineur, ou encore le renforcement des sanctions en cas d'actes de maltraitance à l'encontre d'animaux domestiques. l'interdiction de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la fourrure constitue également une avancée pertinente. Nous ne pouvons toutefois que regretter certains reculs actés lors de l'examen du texte en commission. Ainsi, le rétablissement d'un délai de huit jours avant que l'animal ne soit considéré comme abandonné en fourrière, la réautorisation de la vente des chats et des chiens en animalerie et la réécriture complexe complexe de l'article 12 sur l'interdiction de la détention d'animaux sauvages par les cirques itinérants sont des retours en arrière par rapport aux ambitions déjà modestes, nous semble-t-il, des auteurs de la proposition de loi. Madame la rapporteure, comme

Toutefois, nous partageons pleinement votre position sur l'article 4, qui rendait obligatoire la stérilisation des chats errants pour les communes et les EPCI. La suppression de cette obligation nous paraît justifiée, car il n'est pas envisageable de faire peser une telle responsabilité sur les élus locaux, surtout s'agissant d'une mesure très difficile à mettre en oeuvre.

qu'aux établissements immatriculés ; ceux-ci ont souvent des capacités logistiques et des compétences humaines bien plus importantes que certaines animaleries situées au coeur de nos centres-villes. C'est pourquoi, animés de cette volonté de faire confiance aux professionnels, tout en sensibilisant les acheteurs pour éviter les achats compulsifs,

sens. Mes chers collègues, face à une proposition de loi initialement pertinente, mais peu ambitieuse, et constatant les reculs actés lors de l'examen en commission, nous nous mobiliserons, au sein de mon groupe, pour améliorer les dispositifs et les outils de lutte contre la maltraitance animale. La parole

s'il convient de ne pas réduire l'animal à un mini-humain, on ne décèle pas moins en lui certains états mentaux et émotionnels proches des nôtres. Les conceptions relatives aux animaux ont certes varié dans l'histoire, mais, au Moyen-Âge déjà, on considérait l'animal comme un sujet un sujet digne de respect, avec lequel nous continuons aujourd'hui de nouer des liens d'interdépendance. Nous savons désormais que le langage n'est pas une une barrière infranchissable entre nous. Les animaux s'expriment, sont capables de jugements moraux. Ils sont présents dans toutes les sociétés humaines, et, aujourd'hui, notre cohabitation devrait être solidaire. L'animal est un être vivant avec sa propre identité. En tant que tel, il nous impose de repenser sa condition et de légiférer à son sujet. La protection des animaux reste largement perfectible : de nouvelles dispositions permettraient de renforcer l'arsenal déjà disponible. La condition animale évoluera non pas seulement par la force du droit, mais aussi grâce à un travail continu sur l'imaginaire, qui, seul dans la durée, influera sur les mentalités et les comportements. Ainsi devrions-nous interdire à terme l'élevage intensif pour prendre en compte la sensibilité reconnue des animaux et leur offrir un cadre de vie meilleur, une vie plus saine, un espace en plein air, en un mot des conditions d'élevage concordant avec leurs impératifs biologiques, ainsi qu'une mort plus douce. Il est temps de reconnaître la souffrance animale

en 1884, « si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destiner à la mort »- j'ajoute : ou à la souffrance -« tous nos semblables qui portent museau et ne diffèrent de nous que par un angle facial moins ouvert, nous n'aurions certainement pas réalisé notre idéal.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, madame la rapporteure, chère Anne Chain-Larché, monsieur le président de la section

le Gouvernement a pris la décision, qui lui revenait, de nous permette d'en débattre aujourd'hui. Madame, monsieur les ministres, nous partageons les objectifs de ce texte. Les souffrances gratuites infligées aux animaux sont insupportables

de la volonté de renforcer, en les amendant, les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer la condition animale, même si, comme certains l'ont dit ici, le problème n'est pas complètement traité. Cette proposition de loi cristallise bien des passions : on le voit sur les réseaux sociaux. Cet élan a des côtés positifs, et cela ne m'étonne guère : la cause animale est aussi affaire d'émotions ; elle a à voir avec ce lien particulier tissé par chacun de nous avec les animaux, avec l'intime conviction que le sort de l'homme et celui du règne animal sont intimement liés. C'est en réalité un enjeu qui

pour comprendre l'efficience des dispositifs proposés. Je veux d'ailleurs remercier tous ces professionnels. Ces rencontres furent parfois magiques, je dois le dire. Pour ma part, je n'ai fait qu'un seul des déplacements réalisés par Mme la rapporteure, mais les rencontres que nous avons faites occasion avec des vétérinaires de la faune sauvage, des soigneurs, des entrepreneurs passionnés étaient presque émouvantes, tant la connaissance intime du monde animal et la volonté farouche de sauvegarder les animaux et leur bien-être étaient ancrées en eux, par ailleurs à une grande humilité. Il me semble que tout le monde ici reconnaît le travail sérieux et constructif de Mme la rapporteure, même si des désaccords peuvent exister çà et là- c'est bien ce qui rend les débats fructueux. Aux côtés des auteurs de la proposition de loi, elle a proposé à la commission des affaires économiques de reprendre à son compte, et même de renforcer, certaines améliorations notables apportées par l'Assemblée nationale.

C'est le cas de certaines dispositions- nous aurons ces débats -sur les delphinariums, les animaleries et même les cirques, qui, en sus de l'intérêt des animaux, ne doivent pas conduire à ériger des barrières étanches entre l'homme et l'animal. Enfin, la responsabilité individuelle doit nous guider. C'est elle qui justifie que l'on sanctionne plus durement les actes de cruauté, les atteintes sexuelles, les abandons, les fraudes. C'est elle aussi qui doit nous conduire à ne pas créer une présomption de maltraitance pour tous les professionnels et tous les particuliers au contact des animaux.

nous concentrer sur l'efficacité de nos décisions, qui ne sont pas, madame, monsieur les ministres, des demi-mesures ou de la timidité, mais des décisions pour les animaux, donc pour les hommes.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, à la lecture du texte dont nous allons débattre, on peut se demander ce qu'est devenue l'ambition initiale, tout à fait bienvenue, des auteurs de la démarche.

Sans minimiser aucunement l'importance de ce qu'il en reste, j'observe qu'il n'est plus question que d'animaux domestiques et de quelques cas particuliers d'animaux de rapport. Pour ce texte, comme pour beaucoup d'autres depuis quelque temps, il s'agit moins de régler sur le fond des problèmes de société que de s'attirer les faveurs électorales de catégories bien segmentées de la population française. Autrement dit, comment éviter de se faire reprocher de n'avoir rien fait sur ce sujet important, en faisant le minimum, sous contrainte pour nous, libres parlementaires en principe, de l'article 45 ? Voilà pour le contexte. Le changement de titre opéré en commission ne change rien à l'affaire ; il faudra reprendre le sujet pour significativement « renforcer les liens entre humains et animaux ». Un beau titre, assurément, évocateur des défis à relever, mais pour un texte très en deçà de cette belle ambition, même si le Sénat a tenté de l'améliorer, je salue ici les travaux de la rapporteure. Il eût pourtant été utile que ce débat nous amène à faire progresser en profondeur notre société sur le statut et la place de l'animal dans sa relation à l'homme. Des présocratiques à aujourd'hui, l'histoire de la philosophie occidentale est jalonnée par l'évolution de la pensée éthique de la relation entre l'homme et l'animal. Une histoire mouvementée, qui n'a pas été consensuelle, mais qui a permis de progresser, même si beaucoup certainement reste à faire. Les travaux de Mme Élisabeth de Fontenay méritent à cet égard d'être connus. Plus récemment, la science a pris dans ce débat une place importante. Permettez-moi de citer les apports tout à fait décisifs de la psychologie animale et de l'éthologie, dont M. Boris Cyrulnik est un éminent représentant. Prendre la dimension de ces faits scientifiques, de ces pensées, de leurs évolutions et de leurs controverses nous semble devoir constituer le préalable d'un débat démocratique et législatif vraiment utile à notre pays. Rien de tel ici, ou très peu ! Pourtant, depuis Charles Darwin et quelques autres, la science nous a fait découvrir les mondes mentaux des animaux. Elle nous a appris que la pensée pouvait exister sans langage, que l'animal pouvait aider, par exemple à des fins thérapeutiques, à développer l'empathie chez l'enfant en difficulté et bien d'autres choses. Sans verser dans la position extrême consistant à mettre strictement sur le même plan juridique l'homme et l'animal, notre législation doit évoluer pour mieux reconnaître chez l'animal une altérité porteuse de sens, une subjectivité, une singularité nécessitant le respect dans le règne du vivant sensible. Pour être à la hauteur des enjeux, il devrait en résulter une évolution de notre code civil. Le couperet de l'article 45 nous l'interdit. Toutefois, madame, monsieur les ministres, il serait pour nous éclairant de savoir si le texte que vous proposez, au périmètre réduit, s'inscrit dans une approche spéciste ou antispéciste. une approche spéciste ou antispéciste. L'intention politique fondamentale du Gouvernement est-elle d'accorder aux animaux ou à certains d'entre eux un statut moral supérieur à celui qui leur est reconnu aujourd'hui dans notre législation ? La question que je pose ici n'est pas anodine. Elle emporte une vision de la société, de ses évolutions possibles et des mesures à concevoir pour les prendre en compte dans l'intérêt général de la Nation. C'est aussi une préoccupation pour beaucoup de Français, qui, j'en suis sûr, nous écoutent

morale en action, de la dignité de l'homme dans son comportement vis-à-vis de l'animal- animal qui, comme cela a été rappelé, est un être vivant, doué de sensibilité, même s'il reste soumis à la réglementation sur les choses. Je dois dire tout d'abord que nous ne sommes pas dupes du « en même temps » que représente ce clin d'oeil à une certaine partie des Français, sensible à la cause animale, au travers d'une proposition de loi tout à fait partielle- j'y reviendrai -, quand, dans le même temps, le Gouvernement prépare des décrets visant à restaurer les chasses traditionnelles, censurées par le Conseil d'État en fonction de la réglementation européenne, autre clin d'oeil évidemment,

plusieurs milliers d'entre eux- 10 000 à 15 000 selon les années -meurent chaque printemps dans le golfe de Gascogne, parce que les mesures relatives à la pêche ne sont pas prises. Nous allons éviter le sujet de l'égorgement sans étourdissement

le texte, tel qu'il nous est soumis, prévoit l'interdiction de vente de tous les animaux en animalerie, alors que, à l'Assemblée nationale, le but était seulement d'interdire la vente des carnivores domestiques, chiens et chats. Enfin, en l'état actuel du texte,

la Commission. Une position équilibrée ne doit pas être une position à mi-chemin entre les attentes des uns et des autres. Ce doit être plutôt une position juste, pesant à leur juste valeur chacun des arguments. Il ne s'agit pas de faire du moyen terme pour trouver de l'équilibre.

modifié certaines de nos façons de voir au cours des dernières décennies, les exemples en sont nombreux. Nous devons maintenant faire évoluer notre façon de voir la condition des animaux. Nous sommes tous allés au cirque quand nous étions enfants et nous l'avons certainement apprécié. Nous n'en sommes en rien coupables, mais nous devons revoir la conception que nous avons de la condition des animaux présentés dans les cirques. Enfin, et pour conclure, seul un gouvernement a les moyens d'une grande loi de mise à jour de la question animale.

Forts des progrès de la science, nous ne pouvons plus ignorer certaines réalités. Oui, l'animal est un être sensible avec lequel nous partageons la capacité de penser et de ressentir, mais aussi de souffrir. Dès lors, il y va de notre dignité d'être humain que de faire usage de notre empathie envers ceux que Jules Michelet appelait « nos frères inférieurs » : sans céder à une sensiblerie excessive qui consisterait à assimiler l'animal à l'homme, nous avons le devoir de les protéger de toute de souffrance évitable. C'est là toute l'essence de la proposition de loi de lutte contre l'abandon et la maltraitance animale que nous avons l'honneur d'examiner aujourd'hui et qui, même si ce n'est pas un grand texte, témoigne de l'évolution des mentalités. Cette évolution est une urgence, alors que la France affiche le sinistre record de championne d'Europe des abandons, et, à ce titre, la création d'un certificat de connaissance des besoins spécifiques des animaux de compagnie et des équidés est une excellente chose. Alors que 69 % de nos concitoyens considèrent que la classe politique n'agit pas suffisamment en faveur des animaux, il est essentiel que nous leur apportions des réponses concrètes. De même, le récent choix du groupe Kering, propriétaire de la marque Yves Saint Laurent, de ne plus utiliser la fourrure dans ses prochaines collections témoigne d'un changement de paradigme sociétal, dont nous devons tenir compte. C'est pourquoi je souhaite tout d'abord saluer les avancées consacrées par la commission des affaires économiques du Sénat, qui a examiné ce texte, ainsi que le travail sérieux et engagé de Mme la rapporteure. Je me félicite d'un certain nombre de mesures adoptées par la commission, à l'image de l'interdiction de l'expédition postale d'animaux domestiques et non domestiques, ainsi que celle des offres du type « satisfait ou remboursé ».

Nous pouvons aussi nous réjouir de la création d'une circonstance aggravante pour les actes de cruauté sur un animal lorsqu'ils sont commis devant un mineur. Enfin, je salue la mise en oeuvre d'un arsenal répressif destiné à venir à bout du fléau de la zoophilie. Au XXI siècle, il est impensable qu'un individu déviant puisse exploiter la vulnérabilité d'un animal pour assouvir ses pulsions délictuelles. À titre personnel, néanmoins, j'aurais souhaité que nous empruntions le chemin ouvert par l'Assemblée nationale et que nous décidions du renoncement progressif- en concertation avec les professionnels, cela va de soi -à la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, conformément à l'avis de nombreux scientifiques. Enfin, je ne pourrais conclure sans évoquer la problématique des euthanasies de convenance pratiquées à la demande du propriétaire, un sujet auquel je consacrerai un amendement. Il est essentiel de supprimer la chape de plomb qui pèse sur les épaules des vétérinaires, en introduisant une procédure collégiale obligatoire destinée à accorder une ultime chance à l'animal. Des mesures de substitution à la mise à mort doivent pouvoir être envisagées en cas d'impossibilité pour le propriétaire de continuer à prendre en charge son animal. Mes chers collègues, les attentes croissantes de la population concernant la défense des animaux ne doivent plus être ignorées. Le Sénat, dont l'ADN est de se faire l'écho de l'attente des Français, s'est emparé du sujet. Mais, en partant toujours d'une éthique de responsabilité, chère à Mme la rapporteure, ma conviction est qu'il faudra aller plus loin sur cette question. Protéger les animaux de la violence et de l'abandon, c'est réaffirmer avec force la richesse de notre humanité. La discussion

de l'espèce, une information sur le budget que peut représenter la garde d'un animal. Les abandons sont un fléau qui touche chaque année 100 000 animaux dans notre pays.

Afin d'y remédier, l'amélioration de l'information de l'acquéreur est primordiale : cette information financière relative à la garde d'un animal est donc indispensable pour que la décision d'acquisition puisse être prise en connaissance de cause.

Les documents à remettre obligatoirement lors de la cession sont pour cela un bon outil, tout comme le certificat proposé ici. Le document d'information existant, qui doit être donné à l'acquéreur lors de toute cession, comprend déjà déjà « une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir. »

d'obtenir le nouveau certificat de connaissance. Elle a opté pour une durée de deux ans, alors que l'Assemblée nationale prévoyait une application immédiate. Nous pouvons comprendre la nécessité d'introduire un délai, pour permettre une bonne et juste application de la loi.

Je l'ai voulu long, car il est probable que les décrets d'application, détaillant le contenu du certificat et, surtout, encadrant la manière dont celui-ci sera délivré, ne paraîtront pas immédiatement. Mon souhait était donc que chacun puisse prendre connaissance de la loi avant d'être mis devant le fait accompli.

En l'occurrence, il y a déjà obligation, lors de toute vente ou cession par une association de protection animale d'un animal de compagnie, de délivrer une attestation de cession qui comprend un certificat d'engagement et un document d'information. Ces documents sont en outre spécifiques à l'animal, et pas seulement à l'espèce.

Cet amendement vise à soumettre les détenteurs actuels d'un animal de compagnie à la signature d'un certificat pour le prochain animal qu'ils achèteront après l'entrée en vigueur de la loi, et cela, donc, même s'ils en détiennent déjà un.

qui est d'application directe en France. Dans ce texte, l'animal de compagnie est défini comme « un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales ». Tout est donc prévu, et un arrêté ne me paraît pas nécessaire.

Toutefois, afin d'intégrer au mieux dans le droit existant cette disposition, dont la portée contribue à la sensibilisation des futurs propriétaires d'animaux de compagnie, cet amendement tend à supprimer l'alinéa 11 de cet article 1, qui confie à un arrêté le soin de préciser la notion d'animal de compagnie. de compagnie. L'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà une telle définition, précisant que l'« on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ». Il ne nous paraît pas nécessaire de créer une nouvelle définition juridique de la notion d'animal de compagnie, dans la mesure où celle-ci est déjà encadrée par le droit positif. L'amendement n° 82 rectifié tend à généraliser les formalités de cession qui s'appliquent aujourd'hui uniquement aux ventes professionnelles, c'est-à-dire en refuge, élevage, animalerie ou par des particuliers éleveurs, à tous les particuliers et aux dons. S'agissant du document d'information, notons tout d'abord que le certificat créé par l'article 1 concernera bien les cessions entre particuliers, y compris les dons. J'ai prévu qu'il reprenne le contenu du document d'information L'amendement est donc satisfait sur ce point. En revanche, je ne souhaite pas généraliser le certificat vétérinaire, ni l'attestation de cession. Prévoir un formalisme démesuré pour des échanges non professionnels risque d'inciter à l'abandon. ailleurs, avons-nous réellement les moyens de contrôler le respect de ces dispositions ? Comment l'État surveillera-t-il que tous les dons d'animaux entre voisins ou membres de la famille sont accompagnés d'une attestation de cession ?

de l'amendement n° 9 de notre collègue Fabien Gay, il me semble utile de maintenir un ciblage sur la primo-acquisition. L'objectif principal est bien de sensibiliser les nouveaux acquéreurs.

En effet, avec l'essor des « nouveaux animaux de compagnie », nous ne parlons plus simplement de chiens et de chats ; nous parlons aussi de reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux rares, etc. Pour appliquer la mesure, comment un vendeur saura-t-il si l'animal est considéré comme étant de compagnie

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à établir la nécessité d'un justificatif de domicile validé pour les carnivores domestiques, afin que le détenteur enregistré dans le fichier national ne puisse être contesté.

en ligne, de s'assurer que seules des personnes majeures détiennent un animal. Cela permet, surtout, de limiter le trafic des chiens. Il sera effectivement plus aisé d'identifier un trafiquant en observant le nombre de chiens enregistrés sur le même domicile il sera de même plus difficile pour un trafiquant d'utiliser un prête-nom pour identifier tous ses chiens et il sera plus facile de répertorier tous les chiens d'un trafiquant lors d'une saisie. Cela permet par ailleurs d'éviter les achats « cadeaux », parce qu'il sera bien difficile de fournir un justificatif de domicile d'une tierce personne à son insu. Cela évite, en partie, l'existence de deux sortes d'animaux, qui encombrent particulièrement les refuges. Les premiers, appelés « pits de cave », sont des chiens d'attaque souvent détenus par des mineurs, sans l'accord de leurs parents.

de coffre », utilisés pour le gardiennage, sont détenus dans des conditions peu scrupuleuses, stockés dans des cages, dans des coffres de voiture, sur des balcons, etc. Ces chiens ont tendance à être utilisés par plusieurs « agents

Je n'ai pas eu connaissance de fraudes importantes à cet égard. En effet, dans les cas de vols et de trafics, les trafiquants ne prennent pas la peine de modifier leurs coordonnées auprès de l'I-CAD avant de revendre illégalement des animaux. Aussi, je ne vois pas ce qu'apporterait un justificatif de domicile dans de

Pour toutes ces raisons, je persiste à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

L'objectif est tout simplement d'étendre la compétence des policiers municipaux et des gardes champêtres à tous les animaux concernés par l'obligation d'identification. Aujourd'hui, ces agents ne peuvent intervenir que pour les chiens et chats.

ces établissements professionnels, la loi donne déjà compétence à de nombreux personnels habilités, comme les agents des douanes, ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), les vétérinaires d'État et les inspecteurs de l'administration.

contrôler les animaux des habitants dans les rues ? Pourraient-elles les verbaliser, au même titre que les policiers ? Ce ne sont pas des agents de service public, et je ne souhaite pas leur confier de tels pouvoirs. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Le scrutin est clos.

Toutefois, il apparaît que cet article est contraire au droit européen issu d'un règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et ses actes secondaires. telle modification engendrerait des incohérences avec ce règlement ; elle s'imposerait aux éleveurs d'animaux de rente ; elle désorganiserait la gestion des fichiers nationaux d'identification et de traçabilité des animaux de rente délégués par espèce à différents organismes privés. Pour l'ensemble de ces raisons, les élus du groupe RDPI proposent la suppression de cet article.

pour traiter de manière automatisée les contraventions à cette partie du code rural. D'ailleurs, les délits prévus par le code sont déjà verbalisés électroniquement. C'est le cas, par exemple, des infractions à l'identification obligatoire des chiens et chats. J'y insiste, dans le

? Aujourd'hui, le droit définit le refuge comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet et, enfin, accueillant et prenant en charge des animaux, soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire. Toute activité répondant à ces critères relève de l'encadrement des refuges. Cet amendement vise à inclure dans les catégories d'animaux accueillis ceux qui sont pris en charge sur décision de l'autorité administrative ou judiciaire, c'est-à-dire les animaux réquisitionnés, confisqués ou retirés à leurs